avait pris une initiative de mettre en place un dispositif de contrôle leur application, le Sénat a d'ailleurs adopté à l'initiative du groupe socialiste et républicain, une modification de son règlement pour consacrer et renforcer les capacités de contrôle de l'application des lois, ce texte déclarées conformes à notre constitution, la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, notamment, a confié au rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi la responsabilité d'assurer le suivi de son application, et ce après la promulgation du texte, cette résolution consacre également l'existence du bilan annuel, nous sommes en train de faire, il semble en effet que la loi votée aux yeux de nos concitoyens qui s'impose à tous ceux qui leur sont parfois aux parlementaires, mais aussi, mais aussi aux citoyens, que c'est un peu incompréhensible entre la loi et l'la mise en exécution de la loi, il à la fois beau. Parfois beaucoup de temps et parfois une non application de la loi, l'exemple des textes santé on est une belle illustration je regardais hier 3 textes depuis le textile de Madame Bachelot Madame Touraine, celui d'aujourd'hui, au moins 10 ans et l'ensemble des décrets dont pas tous été pris, je me permets de le dire et compris. Sur un certain nombre de textes, je crois que c'est une illustration, je vais donner maintenant immédiatement la parole la présidente de la délégation du bureau en charge du travail parlementaire et pour nous présenter le le bilan de l'année parlementaire 2017, 2018 41 lois votées lors de cette première session de la législature et je le remercie pour la qualité de son rapport d'information sur le bilan de l'application des lois au 31 mars 2019, madame la présidente. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, depuis près de 50 ans, le Sénat s'attachent à vérifier que les textes réglementaires prévus par le législateur soit pris en temps et en heure, ce travail est le fruit d'un suivi minutieux de chaque commission pour les lois relevant de son ressort, il est également le résultat d'un dialogue de qualité avec les administrations et le secrétariat général du gouvernement, que je tiens à souligner. Le bilan que je vous présente ce matin portent sur les lois adoptées lors de la session 2017, 2018 à la date du 31 mars 2019 sur les 41 loi adoptée, monsieur le président, lors de cette session hors conventions internationales 28 nécessité la prise de mesures d'application, le taux d'application de cette année est de 78 pourcent et même de 86 pourcent si on y exclut les mesures demandées par des articles dont l'entrée en vigueur est différé je souhaite insister sur le fait qu'il s'agit du plus haut niveau atteint depuis que le Sénat procède à cet exercice, pour mémoire, il était de 65 pourcent en 2014 et de 73 pourcent l'année dernière. Cette progression témoigne de la volonté commune du Sénat et du gouvernement d'une bonne application de la loi et de l'utilité de notre exercice annuel tous types de textes réglementaires inclut ce sont ainsi 453 mesures qui ont été prises sur les 589 attendu permettez-moi cependant d'exprimer un 1er regret : le gouvernement ne comptabilise dans ces chiffres que les décrets à l'exclusion des arrêtés, or certaines lois demande la prise d'arrêter et ce chiffre n'était pas négligeable pour la session 2017, 2018 un peu plus de 90 arrêtés étaient attendus, soit 15 pourcent des mesures. J'en viens maintenant au délai moyen de prise des textes réglementaires d'application, là aussi, des progrès ont été faits, les décrets pris le en moyenne en 4 mois et 17 jours ce délai particulièrement court en raison du processus d'élaboration concertation réunion interministérielle consultation et avis obligatoire d'organismes notification à la Commission européenne, passage en Conseil d'État, le cas échéant, 84 pourcent des mesures d'application prises l'ont été cette année dans un délai inférieur à 6 mois, témoignant de la pleine mobilisation du gouvernement pour l'adoption de ces mesures toutefois une moyenne cache toujours de fortes disparités. 11 mesures d'application de loi votées lors de la session 2017, 2018 ont été prises avec un délai supérieur à un an de manière symptomatique de décrets ont été pris en décembre 2018 pour une loi votée en 2010 et ceci sous la pression d'une sanction de la part du Conseil d'État. Ces délais excessifs sont d'autant plus difficile, est difficile à accepter que la loi est votée, de plus en plus rapidement, en 3 ans, le délai moyen de vote de la loi, a diminué de 2 mois et 8 jours, ce délai de vote et de 177 jours je relève qu'à ce titre que la procédure accélérée est devenue la procédure privilégié du vote de la loi, elles représentent 83 pourcent des lois votées lors de la session 2017, 2018 hors conventions internationales, vous comprendrez, monsieur le ministre, notre étonnement lorsqu'il vous faut plus de temps pour rédiger un décret qu'il nous en faut pour voter la loi, je rappelle à cette occasion, la proposition du groupe de travail du Sénat, mis en place dans la perspective de la révision constitutionnelle de créer un contrôle juridictionnel en permettant aux présidents des 2 assemblées, ainsi qu'un qu'à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil d'État, en l'absence de publication des mesures réglementaires d'application d'une loi dans un délai raisonnable, j'en viens maintenant à nos points de vigilance, voire d'insatisfaction tout d'abord, et je pèse mes mots, le taux de remise des rapports de l'article 67 reste désespérément faible seuls 10 rapport sur les vingt-huit loi votées lors de la session 2017, 2018 et nécessitant des mesures d'application ont été déposées, certains sont remis avec un retard très important : le rapport relatif à la mise en application de la loi dite MAPTAM a été remis 48 mois après sa promulgation, perdant ainsi une grande partie de son intérêt, or il ne me semble pas que la rédaction de ce rapport présente une difficulté particulière, en effet, ce document mentionne seulement les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi ainsi que le cas échéant les dispositions de celle-ci, qui n'ont pas fait l'objet de textes d'application nécessaires et on indique les motifs plus encore, il doit nous permettre de comprendre pourquoi telle ou telle mesure n'a pas été prise, bien souvent, les raisons sont légitimes problèmes juridiques négociations en cours avec les acteurs concernés, textes en cours d'examen dans le cadre d'une consultation obligatoire avis négatifs ou réservés du Conseil d'État sur une première version du texte, il s'agit au final des informations que nous vous demandons, dans le cadre du bilan annuel d'application des lois, en outre, le taux de remise des aide des rapports demandés au gouvernement et dont l'échéance est passé et peu élevé, il est à peine de 54 ces non-transmission concernent parfois des rapports que le gouvernement a lui-même demandé, les rapports sont souvent remis avec retard pour 85 pourcent d'entre eux, or les rapports participe à la bonne information des parlementaires mes collègues vous feront certainement par de leurs griefs sur ce sujet, je ne prendrai qu'un exemple, l'article 32 de la loi allure prévoit un rapport concernant le statut unique pour les établissements et services de la veille sociale de l'hébergement et de l'accompagnement, il est depuis le début de l'année 2017 en attente de transmission au Parlement, je note toutefois que 3 rapports nous ont été remis depuis notre réunion avec le secrétaire général du gouvernement à la mi-mai, j'y vois un signe de lutte il stimulation que constitue cet exercice annuel du contrôle de l'application de la loi, nous le savons tous, chacun d'entre nous a pu être tenté de demander un rapport afin de contourner une irrecevabilité financière, il me semble que nous devons collectivement utiliser cet outil à bon escient, permettre l'obtention d'informations utiles au Parlement pour légiférer, évaluer les politiques publiques et contrôler l'action du gouvernement, d'ailleurs, je souhaite rappeler que le Sénat est beaucoup plus strictes depuis quelques années sur les demandes de rapport si nous devons poursuivre notre effort, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que dans ces conditions, nous attachons beaucoup d'importance à la remise des rapports demandés, j'en viens maintenant aux ordonnances, je suis sûr que mes collègues nous interrogerons également à ce sujet, comme l'année dernière, l'argument de la célérité est à relativiser, puisque le délai moyen pour prendre l'ordonnance, une fois la loi donnant l'habilitation promulguée et de 455 jours seuls 3 ordonnances ont été prises dans un délai inférieur à 177 jours qui le délai moyen de vote de la loi, le délai constaté entre la date de demandes de l'habilitation et la prise de l'ordonnance est en moyenne de 727 jours, on peut regretter que les consultations ne se fasse pas ou trop peu, en amont de la demande de l'habilitation, cela permettrait d'une part, d'accélérer la prise des ordonnances, mais surtout cela permettrait au gouvernement de donner au moment où il sollicite l'habilitation, les grands axes, issu de la concertation, nous gagnerions en efficience, mais aussi en transparence, de plus il y a l'importance du nombre d'ordonnances et les sujets traités par celle-ci, qui sont à prendre en considération, on peut tout à fait imaginer que pour des raisons d'agenda législatif tout ne puisse pas rentrer dans l'ordre du jour, il y a peut-être à identifier et à hiérarchiser les sujets pour garder en projet de loi les thèmes majeurs et qui relèverait normalement d'un débat avec le Parlement, je regrette que la ratification des ordonnances se fassent souvent par amendement au détour d'un véhicule législatif cela limite le débat parlementaire et je ne peux me satisfaire de l'argument de l'embouteillage de l'ordre du jour, dans la mesure où le gouvernement détermine au moins la moitié de celui-ci, mes collègues vont certainement vous interroger aussi sur des mesures prévues par des lois relevant de leur compétence à cet égard, votre prédécesseur avait lors du débat de l'année dernière, pris un certain nombre d'engagements, c'est le rôle du Parlement, de vérifier que ces derniers ont été respectées, j'ai donc procéder à un droit de suite sur ces points mis en avant par mes collègues président pour leur importance particulière leur sensibilité ou la récurrence du problème évoqué si dans de nombreux cas, les textes d'application ont été pris plusieurs mesures mises en avant sont toujours attendus, j'en évoquerais une, la liste des États non coopératifs pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, cette liste doit normalement être actualisé tous les ans, or la dernière version date de 2016 lors du débat de l'année dernière, votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait indiqué que cette liste sera actualisée sur la base de l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, alors en cours d'examen mais 6 mois après l'adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude, la liste n'a pas été mise en à jour alors même que votre prédécesseur avait indiqué qu'il faudrait après adoption de la loi procéder à cette actualisation le plus vite possible, nous serons donc très vigilants, monsieur le Ministre aux engagements que vous allez prendre, aujourd'hui, je vous remercie. Merci madame la présidente, il y a quelque chose à méditer l'ordonnance 455 jours. Je rappelle que le principe de l'ordonnance d'un côté, il y a complexité mais il y a aussi celles Alors il faut qu'on se dise où ça sert à rien, ce qu'on fait. Ou alors on se dit que ça n'est plus acceptable dans l'État, je le dis clairement parce que nous voyons la multiplication de ce genre de Lens qui est une manière de contourner le Parlement, et quand on est à 455 jours on peut se dire que on a oublié la célérité comme 1er, facteur d'ordonnance permet ce commentaire parce que il y a un moment, on va pas se réunir annuellement pour constater qu'on est passé de 455 à 452 plus à 470 je me permets de le dire parce que je crois que c'est aussi le respect des équilibres avec le Parlement et en ces temps de recherche d'équilibre, je crois que c'est important, monsieur le ministre. monsieur le président, madame la présidente Leuthard mesdames et messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier d'avoir maquillé, pour la première fois pour cet exercice annuel de bilan et dialogue

c'est inutile stimulation comme vient de le dire, la présidente Leuthard à l'instant, je tiens donc à remercier Madame Valérie Létard, l'ensemble des présidents de commission ainsi que les services du Sénat pour le travail de recensement, sur la base duquel nous allons échanger, je me félicite du satisfecit et cerné au gouvernement par la présidente Leuthard dans son propos liminaire, c'est un travail considérable qui a été réalisé par les administrations sur l'impulsion des ministres et grâce à la coordination du et du secrétaire général du gouvernement, qui nous permet aujourd'hui d'afficher, comme vous l'avez rappelé un taux d'application de la loi de 85 pourcent c'est 10 points de plus que l'an passé, j'ajoute que quatre plus de 90 pourcent des textes sont pris dans un délai inférieur à 6 mois, le taux d'application des projets de loi, celui des propositions de loi et proche de 80 et 85 pourcent, alors même que, par définition, le gouvernement ne peut anticiper l'écriture des mesures d'application des initiatives parlementaires, comme il le fait de le stade de la préparation des projets de loi, j'en viens maintenant au sujet d'insatisfaction exprimée par la présidente Leuthard le 1er concerne concerne les rapports du gouvernement au Parlement, le taux de dépôt des rapports article 67 et de 45 pourcent au 31 mars 2019, s'il est en augmentation par rapport aux années précédentes, au cours de laquelle il avait atteint environ 40 il demeure très insuffisant et n'atteint pas les taux enregistrés au cours des années précédentes 48 pourcent 2017 49 en 2016, 48 en 2015 pour rappeler les chiffres, le constat est également satisfaisant jonchage changeant, s'agissant des rapports ad hoc, dont la production est prévue par le législateur, même le tard l'a dit, on a pu constater par le passé un certain nombre de dévoiement de ces demandes de rapport qui constitue parfois le moyen de contourner une irrecevabilité financière, il s'agit d'un amendement d'appel qui permet d'ouvrir le débat sur un sujet plus que d'obtenir des informations détaillées ou un état des lieux de telle ou telle sujet aux problématiques je partage donc le constat que vous avez fait sur le fait que cette pratique tend à être contenue et que les commissions à l'Assemblée nationale comme au Sénat, encourager une pratique plus parcimonieuse des demandes de rapport au gouvernement, cela renforce dès lors l'exigence qui pèsent sur lui d'y répondre, s'agissant des ordonnances madame Leuthard et le président Larcher à l'instant invite à relativiser l'argument de la sécurité qui il est vrai, parfois utilisé pour justifier d'y avoir recours, je rappelle qu'il est parfois à bon escient par exemple avec l'adoption, le 22 septembre 2017 des 5 ordonnances prises sur le fondement de la loi pour le renforcement du dialogue social, promulguée le 15 septembre 2017, mais l'urgence n'est pas le seul critère qui conduit à privilégier le recours à l'ordonnance le dialogue social et consultations préalable obligatoire mais aussi la notification préalable à la Commission européenne de certaines dispositions ailier dispositions liées au service, en particulier sur Internet ou la définition des caractéristiques de certaines machines ou engins et au respect du délai du stand Style qui s'ensuit, sont autant d'éléments qui font obstacle à ce que la discussion parlementaire puisse avoir lieu au moment même du vote de la loi d'habilitation de même l'agenda parlementaire ne permet pas toujours d'inclure dans des débats, des dispositions d'ordre technique souvent produites pour la transposition des directives européennes pour procéder à de la codification à droit constant, l'ordonnance et donc un élément de gestion du temps normatif et je j'ai entendu tous les éléments d'que vous avez soulevé les uns et les autres au demeurant la comparaison de l'activité législative du Parlement avec le nombre d'ordonnances démontre bien que l'Assemblée nationale et le Sénat ne pourrait délibéré de la totalité de ses dispositions durant la session parlementaire en effet de 2012 à 2018 pour 346 vous voter 350 ordonnances ont été publiées cet élément de souplesse de sous le contrôle du Parlement est défini évoque le chant et parfois même la durée de l'habilitation des ratifie l'ordonnance après qu'elle été prise, il peut alors modifier un texte qui lui paraîtrait pas conforme à son intention initiale,

les critères régissant la liste française ont été modifiés récemment par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude aux critères de l'effectivité de l'échange de renseignements avec la France, a été ajouté celui de la présence sur la liste des pays et territoires non coopératifs de l'Union européenne, la France est un des P. 1er pays qui, conformément aux recommandations du Conseil de l'Union européenne est susceptible d'appliquer des contre-mesures à la suite d'une inscription sur cette dernière liste, nous sommes donc tributaire et dans l'attente de la stabilisation de la liste noire européenne avant d'actualiser la liste française mais le gouvernement, par ma voix s'engage à une mise à jour très prochaine je vous remercie. vous remercie. Nous allons maintenant procéder au débat interactif, chaque orateur. Je peux intervenir pour 2 minutes maximum et gouvernement lui répondra pour une durée équivalente, mais à chaque fois, donc la parole est que représentants des commissions tout d'abord, la parole est à madame la présidente de la commission des affaires économiques Madame Sophie Primas pour 2 minutes. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues sur la commission des affaires économiques, nous ne pouvons pas nous plaindre puisque la moyenne des taux d'application des lois, suivi par la Commission s'établit autour de 90 pourcent donc au-dessus de ce que je vais entendre globalement ce qui apparaît satisfaisant, mais l'analyse des statistiques relèvent quelques surprises et la loi allure par exemple, qui faisait partie du Champ de notre investigation a par exemple vu son taux d'application brusquement augmenté grâce à la suite de la grâce à pardon la promulgation de la loi élan puisque 17 mesures d'application de la garantie universelle des loyers de la loi de la loi allure sont devenues sans objet, sans jamais avoir été appliqué en pratique, vous voyez bien que l'application des lois un problème quand même aussi politique, je voudrais évoquer le sujet comme le président du recours aux ordonnances à travers un exemple, l'article 12 de la loi hydrocarbures qui a été votée le 30 décembre 2007 habilité le gouvernement à légiférer par ordonnances d'ici au 30 décembre 2018 sur 3 sujets, notamment l'extension du mécanisme d'interruptibilité à des clients raccordés au réseau de distribution et le fait de rendre optionnelle, la compensation financière versée aux consommateurs finaux à à force est de constater que la seule ordonnance paru sur le fondement de cette habilitation ne comporte pas ces 2 derniers points le fait que le gouvernement ne fasse pas usage des habilitations, qui l'a pourtant demandé conforte notre commission dans le contrôle très vigilant qu'elle exerce sur l'opportunité du recours aux ordonnances et elle continuera à chaque fois qu'il est possible à leur préféré, monsieur le Ministre, une législation Direct et, à défaut, à encadrer strictement les délais comme le Champ d'habilitation, monsieur le Ministre, nous entendons régulièrement des remarques sur le temps parlementaire et sa lenteur, le délai pour le vote d'une loi serait trop long, alors que la procédure accélérée désormais devenu la norme, il faut cependant reconnaître manière parallèle que le recours aux 2 aux ordonnances ne rime pas toujours nié avec rapidité ni avec efficacité, ni même avec respect de la chose, voter, d'où notre incitation à être extrêmement prudents. Oui, monsieur le président, madame la présidente, Prima sur les ordonnances, j'ai déjà apporté quelques précisions sur les circonstances de lesquelles le gouvernement a été conduit à solliciter une demande d'habilitation, l'argument de leur j'urgence c'est parfois invoquée, je cite un exemple récent qui attestent que parfois, il est juste, mais parfois il ne l'est pas, je le dis bien volontiers d'autres contraintes rend également la demande d'habilitation indispensable comme je l'ai rappelé pour en venir au cas concrets que vous avez évoquée, je viens d'abord sur les hydrocarbures, elle habilité en effet le groupe en effet le gouvernement à prendre des mesures relatives à la contractualisation de capacités interruptibles l'ordonnance est devenue inutile car lors des discussions parlementaires, la modification des articles L. 431 six tiré de et L. 431 6 3 du code de l'énergie a produit les mêmes effets que le Champ de l'habilitation, voilà pourquoi l'ordonnance n'a pas été prises s'agissant de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, enfin à la citoyenneté, vous en avez dit juste un mot pour dire que le gouvernement a autorisé à légiférer par ordonnance sur un délai 2 ans pour 2 sujets pour pour codifier procéder à une nouvelle rédaction de l'ordonnance n'a pas été publié l'habilitation pour procéder à cette nouvelle rédaction du livre 4 la construction qui portent sur les HLM, est intervenu à quelques semaines des élections présidentielles, voilà les éléments que je pouvais vous. Parole Parole est maintenant au président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, Christian Cambon. Merci monsieur le président, la commission des affaires étrangères et de la Défense est globalement satisfaite des taux de ses taux d'application, néanmoins je voudrais faire 3 remarques tout d'abord les rapports que nous demandons au gouvernement sont absolument indispensables à notre travail de contrôle et du reste les exploitons pleinement, c'est ainsi que le rapport d'avril 2019 sur le rythme de livraison des équipements militaires que nous avions réclamé à grands cris et que nous avons fini par obtenir nous a montré, comme par hasard, un retard de livraison des blindés Griffon sur lequel du reste nous allons interroger et la ministre des armées et les industriels dès la semaine prochaine, tout le monde comprend bien que pour exercer un bon contrôle faut être bien informé ma 2ème observation vise à rappeler une nouvelle fois le regret qui est le nôtre, de voir le gouvernement ne pas respecter son obligation de présenter un rapport relatif au bilan politique et financier des OPEX des opérations extérieures, je rappelle qu'il s'agit de la bagatelle d'un milliard 100 millions qui sont dépensés, hein, et que nous voyons chaque jour le prix qui est payé par nos armées, que par ailleurs la situation au Mali et dans tous ces pays se dégrader et donc la moindre des choses serait que le gouvernement respecte cet engagement, nous avons déjà regretté qu'il n'y ait pas de débat sur ces opérations et donc je reformule la même demande, Monsieur le Ministre, pour obtenir un bilan politique et financier des opérations extérieures, enfin ma 3ème observation VISA à peu attirer votre attention sur un cas particulier d'application de la loi de programmation militaire plus directement de sa non-application, en effet, une disposition introduite par le Sénat et qui tendait à rendre plus Agile, les procédures d'achat de certains équipements militaires a comme par hasard été supprimée par le gouvernement lors de sa codification par ordonnance dans le code de la commande publique, alors je vois bien les mêmes motivations du gouvernement, elles sont d'ordre juridique, la rédaction du Conseil d'État serait sans doute plus lisible que les amendements du Sénat je rapproche cela de l'opposition forte que le gouvernement avait manifesté lors de l'adoption de cet amendement et donc on a, on a un peu l'impression qu'il se satisfait, comme par hasard, de la rédaction du Conseil d'État, je ne sache pas que la Constitution donne au Conseil d'État, le rôle de chambre d'appel au débat parlementaire alors néanmoins cette ces observations ont eu tout de même un effet puisque comme pas, nous avons obtenu une vaste réforme des procédures d'achat d'achat qui a été engagé par instructions ministérielles, mais il serait souhaitable que ça ne se reproduise pas, et nous vous donnons rendez-vous à la ratification de cette ordonnance car nous ne lâcherons pas sur ce sujet, je voulais donc attirer l'attention du mini-sur ces points. Au Monsieur Cambon, monsieur le Ministre, ne doutez pas. Je ne doute pas que le président comme ne lâcherait pas. Monsieur le président, Monsieur le Président, quand bon le Conseil d'État, vous venez de le rappeler lors des travaux d'examen du code de la commande publique, a validé l'abandon des précisions introduite à l'occasion du vote de la LPM, il a considéré que le retour à cette rédaction n'excédaient pas le Champ de l'habilitation dès lors qu'il s'agissait de revenir sur la rédaction exact des directives, surtout, il a estimé que cette solution était la mieux à même d'éviter une interprétation trop restrictive des exclusions autorisé pour ces marchés très spécifique, le Conseil d'État ainsi pleinement validé la position du gouvernement consistant à considérer que les illustrations inséré dans le texte de l'ordonnance n'apportait pas de plus-values été contrairement à l'objectif poursuivi plutôt de nature à encourager une lecture restrictive de la disposition en cause une telle lecture a contrario était en contradiction effectivement avec l'objectif poursuivi par le Sénat qui était plutôt de laisser plus de marge de manoeuvre aux acheteurs du ministère des armées, notamment pour les achats supposant une certaine rapidité une grande confidentialité enfin conformément aux engagements pris devant le Parlement lors de l'examen de la LPM, la ministre des armées a pris plusieurs initiatives visant à fluidifier les achats d'une part par une instruction du 28 janvier 2019 relatifs à la politique d'achat du ministère des Armées, la ministre a donné des consignes très précises au service acheteurs du ministère, ceux-ci disposent désormais d'instructions précises les astreignant exploiter pleinement les marges de manoeuvre offertes par les directives européennes, notamment en dominant rend pas le Champ d'application et les souplesses offertes par le recours aux marchés dits exclus, d'autre part, la direction des affaires juridiques et la direction générale pour l'armement termineront fin juin à la rédaction d'un projet décret visant à mettre fin à l'ensemble des sur-transpositions en matière de marchés de défense et de sécurité à simplifier autant que le permet le droit européen, les procédures d'acquisition, la ministre des armées a donc pleinement repris à son compte l'esprit des mesures souhaitées par le groupe parlementaire et en l'occurrence par le Sénat,

Monsieur le ministre, la parole est maintenant René-Paul Savary oui, président de la commission des affaires sociales pour cette commission. Oui merci monsieur le prési dent donc au nom du du président Alain Milon et de la Commission, je voudrais interroger le gouvernement sur ses intentions en matière d'assurance chômage, cette assurance à travers l'application de 3 textes qui sont les lois de financement de sécurité sociale 2018, 2019, et bien sûr la loi pour la liberté d'choisir son avenir professionnel, c'est loin de financement modifier en profondeur le financement de l'assurance chômage pour substituer aux contributions salariale, une part de CSG, je rappelle que le Conseil constitutionnel n'avait admis la présence de ces dispositions dans un projet de loi de financement de sécurité sociale, sa décision du 21 décembre 2017 et que dans les circonstances particulières de l'espèce, considérant que, si les dispositions relatives aux contributions sociales d'assurance-chômage sont étrangères au domaine de la loi de financement de la Sécurité sociale, le législateur a entendu procéder à une réforme en constituant consistant parlant à diminuer les cotisations sociales des actifs, la suite de ces réformes d'ensemble nous a été annoncé par un amendement du coup ouvertement in-extremis. Sur ce projet de loi de liberté de choisir son avenir professionnel et cet amendement, qui est devenu l'article 56 de la loi, il prévoyait une remise en cause de la convention d'assurance chômage pourtant conclut quelques mois plus tôt, et une nouvelle procédure de négociations avec une lettre de cadrage le texte ouvrait par ailleurs le droit à l'assurance chômage pour les démissionnaires et les travailleurs indépendants, ces nouvelles négociations comme chacun sait, n'a pas abouti et il appartient désormais au gouvernement de présenter ses propositions donc ma question est : claire quelle sera donc la traduction donnée par le gouvernement à l'article 56 de la loi pour la liberté, choisir son avenir professionnel est également dans quel calendrier. Je calendrier. Je ministre. Monsieur le président, monsieur le vice-président Savary. Pour tout vous dire, je crains de ne pouvoir vous apporter à l'heure où je vous parle d'une réponse satisfaisante, vous avez rappelé l'historique, sur la réforme de l'assurance chômage, à la suite de l'échec des négociations entre partenaires sociaux et le gouvernement en fait reprise en main le dossier de l'assurance chômage, avec 2 objectifs : lutter contre la précarité et assez inciter au retour à l'emploi. Muriel Pénicaud engagé très large consultation auprès des différents acteurs du marché du travail, les résultats de ces consultations et les décisions prises par le goût d'un gouvernement vont faire l'objet d'annonces par le 1er ministre dans les heures les aider, pour vous donner des éléments de calendrier et vous comprendrez qu'à ce stade, malheureusement je ne putsch dans les heures, ça pourrait être cet après-midi, oui. Vous comprendrez dans ce contexte que je ne puisse pas anticiper sur ces annonces. Bon, donc vous êtes invité à la patience Monsieur Savary. La parole à la présidente de la commission de la culture, de l'éducation, de la Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, au cours de la session écoulée, plusieurs lois ont été prévenus le dans les secteurs de compétence de la commission de la la culture notamment 3 qui concernent les domaines de l'enseignement supérieur et de l'enseignement scolaire, je concentrerai mes questions sur celle-ci, 2 d'entre elles, je le rappelle était d'origine parlementaire, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat dont notre collègue Françoise Gatel était initiative et la loi relative à l'encadrement de l'utilisation des téléphones du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire proposée par nos collègues députés le 3ème texte était d'origine gouvernementale, il s'agit de la loi d'orientation et de réussite des étudiants sur ces 3 textes, 2 d'entre eux nécessité je m'attarderai pas sur la loi dite elle puisqu'elle a fait l'objet d'un travail de mise en application rapide et complet, ce dont nous pouvons nous féliciter, je voudrais pas qu'on ne m'a m'appesantir sur la loi, or, nous les premiers décrets, arrêtés sont parus le 9 mars 2018 jours de la publication

et ce, à quelques jours de la date limite fixée aux lycéens pour formuler leurs voeux d'après nos calculs, cette loi est à présent aux 3 applicable, mais il y a des mesures manquante à ce jour, et notamment de dispositions qui revêtent une importance particulière à nos yeux, car elles ont été introduites par notre assemblée, même à l'occasion de l'examen du texte, il s'agit d'une part, du fonctionnement et de l'organisation de l'Observatoire national de l'insertion professionnelle que nous avons créé à l'article 7 du texte et son fonctionnement et son organisation n'ont toujours pas été précisées par arrêté pourtant cet observatoire serait important il serait chargé de produire des statistiques sur l'insertion professionnelle des étudiants afin de guider ces derniers dans leur choix d'orientation, d'autre part le cas national fixant les conditions de scolarité d'assiduité applicable aux étudiants introduit à l'article 10 n'a fait l'objet d'aucune mesure réglementaire, aussi je me tourne vers le ministre pour lui demander si le gouvernement envisage de donner à ces 2 dispositions pour nous importante, une tradition concrètes rapidement dans les semaines à venir. Le ministre. C'est le président, madame la présidente Morin-Desailly mauvais interrogé en particulier sur la loi dite loi, or les cette mesure voyant des décrets ont été appliquées dans un délai moyen de 3 mois permettant d'un tenir d'obtenir

l'arrêté de création de cet organisme est en cours de finalisation et devraient pouvoir être publiée pour répondre précisément à l'horizon de la fin de l'année 2019 à la faveur d'une discussion en cours avec les universités sur le fonctionnement de ce nouveau dispositif est la représentation des établissements en son sein, en pratique, s'agissant du 1er cycle et données propres à l'insertion professionnelle de chaque formation se sont déjà renseignés sur Parcoursup sur les quatre Muttenz 1500 formations présentes la finalité de cet observatoire sera ainsi de mesurer à l'horizon de la montée en puissance de Parcoursup les évolutions en cours en matière d'insertion professionnelle, les premiers résultats sont donc on tonnes attendue pour la fin de l'année universitaire 2020, c'est-à-dire une fois que les premières cohortes d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur via Parcoursup auront atteint le niveau L3 ou autre, assure l'obtention de leur BTS ou de leur DUT, l'autre arrêté concerne le cadre national fixant les conditions de scolarité d'assiduité applicable aux étudiants, ce texte fait actuellement l'objet d'une concertation avec les organisations étudiantes et les universités, le texte de l'arrêté devrait être ainsi pouvoir édicter dans les toutes prochaines semaines avant la rentrée prochaine dans la mesure du possible, il s'agit d'un sujet sensible, il fallait prendre le temps de la concertation. La parole est maintenant au président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable que Hervé Maurey et vous avez la parole. Merci monsieur le président, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme chaque année, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a malheureusement constaté un taux encore insuffisant d'application des lois relevant de son Champ de compétences, aussi bien pour les décrets, seulement 60 pourcent des décrets concernant la loi ferroviaire voté il y a un an, ont été publiés que pour la remise des rapports à peine l'amour à peine la moitié des rapports demandés au gouvernement sont rendus en moyenne je souhaiterais cette année évoquer plus précisément le fait que le gouvernement recours aux ordonnances de plus en plus souvent et sur des sujets de plus en plus important, comme nous avons pu le constater là aussi sur le projet de de loi ferroviaire sur le pacte ferroviaire, or, à l'occasion d'échange récent avec le Conseil d'État, nous avons évoqué le fait que le gouvernement ne savait pas toujours lui-même quel périmètre en terme d'habilitation lui serait utile au moment du vote de l'habilitation. Cela conduit au fait que dans certains cas des habilitations, ne sont pas toujours suivies d'ordonnance et que dans d'autres cas des ordonnances excède le périmètre de l'habilitation consentis par le Parlement, cette situation est d'autant plus regrettable que le Parlement est fréquemment contraint de ratifier les ordonnances, au détour d'amendements, disons, j'ai donc 3 questions à vous poser monsieur mise sur ce sujet est ce qu'il y a une réflexion menée au niveau interministériel sur l'opportunité de recourir aux ordonnances et surtout sur le fait qu'on y recourent de plus en plus fréquemment pour réduire artificiellement la taille de textes et obtenir une inscription d'un projet de loi à l'ordre du jour, c'est ce qui était le cas pour la version 1 du projet de loi ceux relatifs à l'économie circulaire peut-il être envisagé 2ème question de rendent les avis du Conseil d'État public en ce qui concerne les projets d'ordonnances et notamment les remarques du Conseil d'État, par rapport à ce Champ d'habilitation lorsqu'il n'est pas respectée 3ème question alors que 4 ordonnances très importantes ont été prises sur le fondement de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire quel véhicule législatif et quel calendrier sont envisagées pour la ratification de ces ordonnances enfin j'aimerais dans les quelques secondes qu'il me reste pas, d'ailleurs vous interpeller sur l'application qualitative des lois puisque dans la Commission nous avons été nombreux à souligner que, malheureusement, très souvent, les décrets, les circulaires ne respectent pas la volonté du législateur et j'aimerais savoir si vous envisagez d'y remédier et si oui comment.

mort et et posé 3 ou 4 questions : je vais essayer de répondre, aussi précisément que possible dans le temps imparti sur le 1er point, j'ai donné des éléments de réponse dans mon propos liminaire sur le recours aux ordonnances pour des raisons parfois technique parfois trop avancé comme des raisons de calendrier d'accélération du calendrier, c'est vrai, ça peut être justifié et ça peut être des éléments qui peuvent être utiles et parfois ça l'a été, pas toujours, je reconnais bien volontiers, vous m'interrogez sur le fait, si le gouvernement entend publier les avis du Conseil d'État sur le projet de loi d'habitat d'habilitation sur les ordonnances, l'idée n'est pas pour le gouvernement de le faire pour bien séparer la question de la législation, d'une part, et la question. Des décrets d'application de l'application des lois, le 3ème sujet que vous évoquez, c'est les 4 ordonnances ferroviaire pour vous répondre plus précisément l'ordonnance de 1018 11 35 du 12 décembre portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services. Le transport ferroviaire de voyageurs, un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement le 27 février 2019 la 2ème. Ordonnance du 2000 1983 du 11 mars 2019 relatives au cas de fixation des redevances liées aux infrastructures, a été déposé devant le Parlement le 29 mai 2019, l'ordonnance du 30 avril 2009 portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sera déposée devant le Parlement, au plus tard le 1er août 2019 enfin l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF un projet de loi de ratification sera déposée devant le Parlement, au plus tard le 3 septembre 2019 le du gouvernement étudiera les modalités ensuite de ratification de ces ordonnances enfin 4ème point sur. L'application qualitative de la loi, c'est l'objet d'ailleurs du travail que nous faisons, ce matin, devant vous, on peut pas en faire si je peux me permettre une généralité, je pense qu'il y a des cas on a un problème d'applicabilité de la loi et puis d'autres qualitatif, ce que vous voulez dire ce que vous vouliez dire je pense mais dans d'autres cas, c'était pas le cas, mais il faut que nous sur le travail avec le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale pour en la loi plus applicable et plus qualitativement applicable. C'est d'ailleurs à des défauts de la procédure accélérée systématique de ne pas pouvoir affiner ce qui rend parfois les votes et inapplicable, enfin des décisions inapplicables, monsieur le président de la commission des finances monsieur et blé. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, pesant punition chaque collègue je l'essentiel après les propos de Valéry, l'état de mes collègues pour m'arrêter sur 3 points précis de préoccupations de la commission des finances, le 1er point concerne l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 2018 pris notre initiative qui prévoyait un dispositif de plafonnement des frais et commissions payées lors de l'acquisition d'un logement, faisant l'objet du dispositif de défiscalisation Pinel ce décret n'est toujours pas pris le secrétaire général du gouvernement nous a indiqué que le retard s'expliquait par la nécessité de consulter encore le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, le ministre de la ville et du logement que nous entendions la semaine dernière a réitéré cet argument cette réunion d'une instance consultative ne devrait pas néanmoins expliqué que 18 mois après le 1er vote du Sénat, les dispositions ne sont toujours pas opérationnels, le gouvernement peut-il donc désormais s'engager sur une date de parution de ce décret, le 2ème point concerne l'article 171 de la loi de finances pour 2018, qui prévoyait de rendre gratuite la circulation sur autoroute pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opérations le MCG nous a répondu que les sociétés concessionnaires doivent se rapprocher des SDIS afin de prévoir dans les conventions, même la prise en charge par ces sociétés de ces frais comptez-vous assurer la pleine mise en oeuvre des mesures ou laissez-vous finalement la main aux sociétés de Kloten in fine et au financement par les départements, car c'est ça que cela signifie enfin nous regrettons que seulement 6 des 16 textes d'application de la loi relative à la lutte contre la fraude, été pris concernant la responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA le ministre Gérald Darmanin s'est engagé en réponse à une question que je lui posais en séance le 29 mai dernier à ce que la mesure d'application soient publiés pour le premier, dont acte, cette même date, peut-elle être tenue pour les autres dispositions du projet de loi comme la publication des sanctions administratives pour les personnes morales, le fameux Neiman et les nouvelles modalités de fonctionnement de la commission des infractions fiscales, suite à la réforme du verrou de Bercy. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le président, Monsieur le Président et blé en ce qui concerne l'application de la loi de finances pour 2018 sur l'article 68, je ne me rappelle pas ce pour quoi le retard a été pris, vous l'avez fait mieux que moi, une réunion interministérielle de validation du projet décret a toutefois été organisée le 19 avril 2019, le Centre national au Conseil national de la transaction la gestion immobilière désormais au complet se prononcera sur le projet relatif au plafonnement des frais le 19 juin prochain, ouvrant la voie à la publication du décret durant l'été 2019 pour vous réponde précisément sur l'article 171 afin de trouver une solution permettant d'assurer la gratuité des péages aux véhicules des pompiers lors d'une intervention une négociation était conduite par le ministère des Transports, avec l'ensemble des sociétés concessionnaires d'autoroutes qui a permis de faire progresser le sujet la gratuité serait traité par des mesures commerciales que les concessionnaires accorderait aux véhicules des indices qui empruntent le réseau autoroutier afin d'intervenir sur des sinistres, quel que soit le lieu de l'intervention je précise sans facturation au conseil départementaux ni compensation financière de la part de l'État, le périmètre de l'accord couvre aujourd'hui 90 pourcent du réseau autoroutier concédé les concessionnaires rendront compte d'ici l'été de l'actualisation des conventions qui les lient au SDIS en ce qui concerne enfin la loi relative à la lutte contre la fraude, le projet d'arrêté sur le paiement solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA a été mis en consultation auprès des professionnels, le 7 juin dernier à la suite de cette consultation qui s'achèvera le 5 juillet le 5 juillet la Commission européenne sera saisie, conformément à la directive européenne de 1035 1535 la durée de cette consultation obligatoire du fait de l'impact du texte sur les services numériques et de 3 mois, dans ces conditions, la publication de l'arrêté interviendra au second semest cependant, à la suite de la consultation des professionnels, le projet d'arrêté devrait stabiliser pour une présentation des modalités de mise en oeuvre aux parlementaires avant l'examen du PLF, quand bien même l'arrêté n'aurait pas encore été publié sur le fonctionnement de la commission des infractions fiscales, le décret 2000 19567 du 7 juin relatifs à la procédure applicable, a été publiée au Journal officiel, donc le 7 juin ce décret s'applique également le dispositif relatif Onem

au 31 mars 2019 91 pourcent, les mesures d'application des lois qui sont passés par la commission des lois, qui représente un échantillon de la moitié des textes législatifs avait été prise le taux l'an dernier était de 72 le 2ème, chose que je peux vous dire c'est que parmi les textes qui ne sont pas pris, il y en a qui sont très importants, j'attire notamment l'attention du gouvernement sur le texte qui est destiné à protéger les sapeurs-pompiers et les surveillants de l'administration pénitentiaire, en leur permettant le recours à des caméras mobiles, les décrets ne sont pas pris et ça fait trop longtemps, la 3ème, chose que je veux vous dire, c'est que les délais pour prendre les décrets sont souvent plus longs que les délais pour voter la loi, alors même que le recours à la procédure accélérée est pratiquement devenu le droit commun, comme le rappelait tout à l'heure, la présidente Valérie Létard, ceci n'est pas normal, nous avons, dans certains cas, des mesures d'application qui prennent 2 ans 12 décrets d'application qui sont sortis dans la période récente porte sur des dispositions législatives qui avaient plus de 2 ans, enfin, et là aussi, je ne serai pas original par rapport à ce que nous a dit tout à l'heure, la vice-présidente, l'État les ordonnances. On nous dit qu'il faut faire des ordonnances pour aller plus vite mais alors le record de lenteur, c'est les ordonnances qu'ils détiennent et nous avons le cas par exemple pour des sujets qui ne sont pas négligeables comme l'immigration, hé bien, nous avons des textes qui, 9 mois après la promulgation de la loi disent après son dépôt ne sont toujours pas pris, enfin il y a quatre mesures d'habilitation pour la loi de programmation pour l'outre- mer, tu vas te 8 février 2017 aucune suite. Alors si nous devons vous habilité, monsieur le ministre, à prendre des ordonnances, nous ne le faisons qu'à regret mais qu'au moins ces dispositions soient prises et quand elles le sont qu'elles le soient suffisamment vite, c'est le voeu que je formule. Que lui, distraire, vous allez répondre aux voeux du président bas. Je vais essayer, monsieur le président, Monsieur le Président, bah je ne reviens pas sur le taux d'application que vous avez évoqués, qui est plutôt pour le coup, un point positif. Concernant la loi relative à l'mais nisation des caméras mobiles le 1er point vous avez évoqué le projet décret concernant l'expérimentation de l'usage des caméras mobiles par les sapeurs-pompiers, a été transmis au Conseil d'État le 31 mai 2019. Son examen par la section de l'Intérieur est prévue le 9 juillet 2019. Le projet décret concernant l'expérimentation l'usage des caméras mobiles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire est en cours de finalisation, ainsi que la doctrine qui fixe le cap de l'expérimentation avant la saisine de la CNIL, puis du Conseil d'État, j'ajoute que la mesure portant application de l'article L 241 tiré 2 du code de la sécurité intérieure, relative à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été appliquée par le décret du 27 février 2019 concernant le recours aux ordonnances, beaucoup de choses ont été exprimées, et vous avez prolongé ce qui avait été exprimée sur les ordonnances. L'argument de la célérité, je le répète, n'est pas le seul qui justifie le recours à l'article 38 de la Constitution, mais je le rappelle, la comparaison l'activité législative du Parlement avec le nombre d'ordonnances voter démontre bien que l'Assemblée nationale et le Sénat ne pourrait délibéré de la totalité des dispositions durant la session parlementaire, ça n'empêche les éléments d'appréciation qu'on on peut partager, que vous avez fait sur les ordonnances sur les 2 exemples d'habilitation, les exemples d'habilitation, vous avez cité et qui figurait dans la loi pour une immigration maîtrisée, le droit d'asile pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, pardon, le gouvernement n'a pas pris les ordonnances correspondantes, mais c'est parce que le terme de l'habilitation respectivement fixées mais on peut aussi en parler effectivement au 9 septembre 2001 pour la. Et au 9 mars 2020 pardon 2020 9 septembre 2020 pour l'un et de MAAF, mars 2020 pour l'autre, enfin j'ai bien noté les remarques que vous avez prise sur l'est de Gap, qu'il y a, si je peux me permettre entre le la la rapidité du vote de la loi et le la la lenteur de la prise des décrets je lui transmettrai l'ensemble des collègues ministres-.

le suivi des résolutions européennes adoptées par le Sénat sur le fondement de l'article 88 K de la Constitution, mérite d'être ici, du rapport d'information que j'ai présenté à ce sujet, pour la 4ème année consécutive, il ressort que le Sénat et vigilant sur les affaires européennes et plutôt entendu à Bruxelles une résolution européenne ont des conséquences directes sur les négociations qui conduisent à l'élaboration de la législation européenne et donc sur la législation française, 2 points méritent d'être soulignée dans plus de la moitié des cas nos résolutions ont été prises totalement ou très largement compte je peux citer celle relative au filtrage des investissements Directs étrangers dans l'Union aux directives de négociations en vue d'accords de libre-échange avec l'Australie et le Nouvelle-Zélande à la cybersécurité en Europe ou encore au détachement des travailleurs, enfin le 2ème point dans plus de 25 pourcent des cas les positions du Sénat ont été partiellement suivie par exemple sur le programme de travail de la commission pour 2018 : la réforme de l'Initiative citoyenne, la convergence sociale dans l'Union européenne ou encore la politique régionale au service de la cohésion sociale, ces 2 points particuliers, reposant également sur le socle européen des droits sociaux dont on mesurera par par la suite l'importance nos résolution constitue l'instrument efficace d'un véritable dialogue avec le pouvoir exécutif, je me félicite de leur est l'amélioration de l'information délivrée par le GE et de la disponibilité du ministre en charge des affaires européennes pour une audition interactif dédié au suivi des résolutions européennes notre commission considère cette audition annuelle comme un moment essentiel du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en matière européenne, enfin, nous sommes très attachés à la procédure permettant à notre commission de formuler des observations sur les projets ou aux propositions de loi contenant des dispositions visant à intégrer en droit national, le droit de l'Union européenne, cette procédure que nous avons utilisées à 5 reprises. Doit permettre de mieux lutter contre la surtransposition qui, en la matière ne favorise pas la compétitivité de notre pays, mais participe par malgré tout à l'harmonisation dans l'espace communautaire. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, Monsieur le Président Vizer, vous avez fait un bilan plutôt positif je crois du travail qui est fait avec l'exécutif sur ces sujets-là, effectivement, on peut encore améliorer les choses, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, sur ces questions-là jour enfin sur les questions de transposition ou de sur-transposition vous vous dire que le gouvernement veille à éviter les phénomènes de surtransposition que nous avons tous ces les uns et les autres, puis parfois regretter à cette fin, le 1er ministre a signé dès le 26 juillet 2017 une circulaire relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leurs impacts, elle a proscrit en principe toute mesure de transposition allant au-delà des exigences minimales d'une directive et a strictement encadré des dérogations susceptibles d'être ménagés. C'est pourquoi, soit nous tous nous suivons avec intérêt le bilan du travail que vous menez au sein de votre commission. Je vais maintenant la parole au représentant des groupes. Tout d'abord, la parole est notre collègue Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur l'application des lois est particulièrement nécessaire en raison à mon sens de la remise en cause croissante de l'action législative que soit d'origine gouvernementale ou parlementaire, cela doit nous interpeller, je pense que l'une des réponses à apporter pour retrouver cette confiance et l'intérêt des Français dans dans la chose publique, se trouve dans l'amélioration de la qualité de la loi et dans la rapidité de son application et les Français attendent du Parlement de rendent la loi plus lisible, plus percutant, plus efficace et surtout plus simple 3 remarques : il faut se donner les moyens de l'effectivité d'une loi avant d'en voter une autre, il faut que le politique résiste à tout prix à la tentation de fabriquer la loi comme simple effet d'annonce, ne faisons pas de la loi, un outil de communication nos politiques publiques souffrent d'un manque de cap clair courageux et réaliste, entraînant souvent un certain nombre de contradictions et incohérences et un exemple assez symptomatique, je sors dans le domaine des politiques publiques environnementales, les Français ont le sentiment que ces grandes lois sur l'environnement depuis la loi de la sur la transition énergétique de 2015 sont inconsistantes, soit les objectifs sont fixés sur le très long terme et nous on ne nous engage pas réellement soit une leçon sur le très court terme et donc irréaliste discréditant ainsi la parole publique l'objectif intenable de 50 pourcent de parts électrique du nucléaire d'ici 2025 on est le meilleur exemple et la programmation pluriannuelle de l'énergie va repousser l'échéance à 2035 et rentrer, ainsi en contradiction avec la loi de 2015, premières victimes de ces incohérences dans les politiques publiques environnementales, c'est l'environnement également, en second lieu, le porte-monnaie des Français, alors Monsieur Münich pour que la loi devienne crédible et efficace, veiller à l'impératif de la cohérence et du réalisme pour davantage aussi de stabilité législative. Je le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, je partage, nous partageons les éléments que vous avez évoquée, vous avez parlé de la nécessité de rétablir la confiance six, les citoyens et la loi et la production de la loi et vous avez tout à fait raison, vous avez évoqué 3 3, la question de de l'effectivité de résister à la tentation de l'urgence ou parfois des effets d'affichage. Et à tenir des caps, c'est ce que nous ayons sur le le sujet que vous évoquez, en particulier sur la transition énergétique, on pourrait revenir d'ailleurs sur des lois, encore hanté, je pense à la loi Grenelle, on a donné des CAP et parfois on a, on a mal expliciter ce que pouvaient être les horizons qui était donnée aux citoyens, y compris dans cette loi, qui avait pourtant un certain nombre de caractères utile la stabilité oui vous reconnaîtrez juge j'imagine, j'espère, enfin, c'est le texte que vous, qui va être soumis aux assemblées sur la loi énergie effectivement, nous avons décidé de reporter de 2025 à 2035 pour des raisons de cohérence et de de mise en pratique concrète de cette loi parce que, reconnaissons que telle qu'elle était posée en 2015 la loi sur la transition énergétique ne permettaient pas de répondre aux objectifs qui étaient assignés. Pour son faire de griefs à à cette loi et à ceux qui l'ont voté, reconnaissons qu'elle, elle posait des termes et des oeufs incantation dont on savait très bien malheureusement parfois à l'avance qu'elle n'était pas, on n'était pas capable de les mettre en oeuvre et donc je je partage votre sentiment, la stabilité, la cohérence, ça permet aussi aux acteurs économiques, de pouvoir se se positionner et effectuer les transitions nécessaires, donc on a besoin de nez la lisibilité aux acteurs pour que les transitions se passe avec un cap qui soient tenu un coq qui soit être crédible et un cap qui soient tenus tenable si je peux dire et c'est à cette cohérence-là qu'on essaie de se tenir, vous avez évoqué ces sujets-là, il y en aurait bien d'autres, mais en particulier sur la quasi-sur la transition énergétique, on a besoin de de tenir les caps que vous avez évoqué, c'est ce qu'on essayera de faire et c'est ce qu'on essaie de faire sur la loi concernant l'énergie sur les autres lois qui relèveront de ce Champ-là. Merci, la parole est Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président, d'abord je vous remercie d'avoir cité eux résolution du notamment à notre collègue Franck Montaugé qui a été validé par le Conseil constitutionnel et qui permettra aux rapporteur de poursuivre leur travail après la promulgation des lois, je voulais demander à monsieur le ministre, si le gouvernement compte s'affranchir de cette habitude néfastes de déposer tous les textes en procédure accélérée, ce qui apparaît d'autant plus étrange que si s'est accéléré c'est urgent et si c'est urgent, ne comprend pas qu'il faille dans ce cas-là plusieurs années pour que les décrets paraissent ensuite je voulais vous appeler votre attention, monsieur le Ministre, sur le fait que, d'après une statistique qui a été faite par les services de la commission des lois 68 pourcent des propositions de loi adoptée par le Sénat reste en instance devant l'Assemblée nationale et comme dans le sens inverse, ça doit être sans doute du même ordre, il y a une grande déperdition de temps législatif, je vais prendre un exemple très concret, nous avons adopté à l'unanimité une proposition de loi sur la plus juste représentation des communes au sein des intercommunalités, il va falloir que cette disposition soit appliquée au moins pour une partie de la proposition de loi. Soit ce soit soit adoptée avant le 1er septembre avant le 30 septembre précisément puisqu'on a reporté d'un mois, et il y a une partie de cette proposition de loi qui émane de Madame Jacqueline Gourault quand elle était sénatrice donc est-ce que vous prendrez les moyens de faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse adopter quelque chose avant cette date, parce que si on n'adopte pas cela avant cette date, hé bien on ne pourra pas

Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Je je reviens d'un mot sur la procédure accélérée, je partage le sentiment parce que c'est une réalité que, désormais, c'est quasiment plus pardonnerez l'expression devenue une procédure de droit commun, reconnaissons aussi qu'elle est une procédure de droit commun, non pas tant seulement depuis ce quinquennat mais d'ores et déjà, le Quai d'État le quinquennat précédent avait largement et parfois avant, fait de la procédure accélérée, une procédure de droit commun pour répondre, pour le reste, vous avez sur les propositions, en particulier le tableau de bord statistique en ligne sur le site du Sénat, entre le 1er octobre et le 26 mai 2019, première étape 2018 et 26 mai 2019 46 textes ont été définitivement adoptés 17 conventions 14 projets de loi et 15 propositions de loi dont six du Sénat l'absence d'obligation pour le gouvernement d'inscrire sur son hôte du jour prioritaire dans une assemblée des propositions de loi adoptée par une autre assemblée n'empêche donc pas les initiatives parlementaires en partie en tout cas de prospérer le gouvernement contribue grandement vous par exemple, parce que les propositions de loi sénatoriale soit inscrite à l'heure du jour de l'Assemblée nationale. Sous réserve de la parution du décret du président de la République, convoquant le Parlement en session extraordinaire à l'Assemblée nationale devrait ainsi à s'être saisi cette année, cet été, pardon de 5 propositions de loi sénatoriale, parmi lesquels la proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles, elle a dit à la diversité et aide à la diversité des territoires, la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse

tout loisir d'inscrire des propositions de loi transmis par l'eau, transmise par l'autre assemblée ainsi que d'ailleurs les groupes d'opposition minoritaire dans le cadre dans l'de leur journée réservées, cela relève aussi du dialogue entre les groupes qui viennent d'eux-mêmes horizons ou pas, j'observe que certains groupes, je ne veux pas dénoncer ici, veille à ce que leur textes puissent poursuivre leur parcours législatif jusqu'à leur terme, dans les 2 assemblées, j'ajoute enfin que les règles de partage de l'Ordre du jour sont souples et que non seulement il arrive au gouvernement d'inscrire des propositions de lois sur son nom 2 jours mais qu'il arrive aussi aux assemblées d'inscrire des projets de loi sur le leur. Merci. Oui, sur les dates. Comme il y a un texte qui va venir qui va essayer de rassembler un certain nombre d'éléments, pardon, président, c'est d'ailleurs, vous m'aviez tendu la perche, si je peux dire, c'est sans doute dans ces textes là, on verra, sous réserve de la production du texte que ces éléments bien, j'ai bien noté les contraintes d'agenda et nous avons bien noté des contraintes d'agenda, sinon que je connais un peu, en septembre, sinon c'est inefficace bien noté, Merci monsieur le président, monsieur le président, Monsieur le Ministre, régulièrement dénoncé l'inflation législative reste néanmoins forte alors même que la procédure, ça a été répété plusieurs fois accélérer devient la règle habituelle de vote de la loi 83 pourcent des lois adoptées l'ont été en urgence en 2017, 2018 contre 77 l'an dernier, cette accélération rend difficile l'application des lois, même s'il faut se féliciter, cela a été dit du fort taux d'application des lois 78 il est cette année encore en augmentation, cela traduit, comme le souligne Valérie Létard dans son excellent rapport la bonne mobilisation du gouvernement sur la question et à travers elle le respect du travail parlementaire, ce qui est toutefois paradoxal, c'est que l'on nous impose en amont la procédure accélérée, mais qu'il faut attendre en aval des mois et des mois, 4 mois et 11 jours exactement pour que ceux qui ont demandé la procédure accélérée publie les textes d'application, c'est au point que la mise en application des lois et parfois la plus longue que leur adoption dont le délai moyen, lui, et qu'en constante diminution, seulement 60 177 jours la session 2017, 2018 soit un délai raccourci de plus de 2 mois en seulement 3 ans, le Parlement légifère rapidement et l'expérimentation du Sénat sur la législation en commission en elle le sait, montre aussi que beaucoup de choses ont été faites à l'initiative du Parlement pour améliorer la capacité à produire de la loi allant fois rapidement et dans de bonnes conditions,

l'un de mes prédécesseurs, Roger Karoutchi, avait dit sa grande expérience que quand on est parlementaire, on veut du temps et qu'on aille de gouvernement, on veut aller plus vite, ce qui est vrai s'agissant du temps parlementaire s'inverse quand on aborde le temps réglementaire, c'est ce que vous avez dit pour un certain nombre d'entre vous, et au-delà de de ces éléments, il arrive que nous aurions à certaines difficultés qui peuvent retarder le présent, la prise d'un décret, le cas de l'application de l'article 68 de LFI pour 2018, qui a été évoqué un peu plus tôt est assez parlant, le décret n'a pu être pris pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, je n'y reviens pas, on peut également se heurter à des difficultés de mise en application pratique ou bien des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire, qui n'avait pas été ou pas pu être anticipé mais vous me permettrez tout de même une certaine. non pas d'autosatisfaction parce que c'est toujours mauvais aloi d'être dans l'autosatisfaction, mais en tout cas de donner des éléments puisque 85 pourcent des décrets d'application d'application sont publiées dans un délai de 6 mois et que le délai moyen de prise des textes d'application. Est en diminution, outre l'organisation régulière de réunions interministérielles pour chaque loi nouvelle le suivi de l'application de la loi fait toujours l'objet de communication conseil Münich effectuerait moi-même une communication le 10 juillet prochain sur ces sujets et nous y veillons scrupuleusement enfin j'organise régulièrement avec le secrétaire général du gouvernement, des comités interministériels de l'application des lois qui rassemble l'ensemble des directeurs de cabinet des membres du gouvernement pour avancer et accélérer les processus cette mobilisation permet ainsi au gouvernement non seulement publier la grande majorité des décrets en temps et en heure, mais aussi de s'assurer d'une application uniforme des textes de loi qui soit d'initiative gouvernementale ou parlementaire, j'ajoute qu'il s'agit d'un effort tout à fait considérable pour certains textes gouvernementaux qui doublent ou triplent de volume à l'issue de l'examen parlementaire puisque par des fans, ici on ne travail d'écriture ne peut commencer en amont, dès le stade de finalisation des dispositions du projet de l'eau. Je le dis au Sénat mais c'est n'est pas forcément au Sénat que cette inflation législative et la plus. Merci, la parole est à notre collègue Alain Richard pour le groupe de la République en marche.

le seul point sur lequel je voudrais souligner, il a indiqué une petite différence, c'est que parfois une loi opère une réforme. Et nous avons quelques expériences, nous rappelons que les réformes sont difficiles dans ce pays et qu'elles sont généralement conflictuel, donc ceci s'entend parfois, même de façon assez sonore pendant le débat législatif mais ça se manifeste aussi ultérieurement dans la phase réglementaire puisque les éléments du conflit sont toujours là et les protagonistes sont toujours aussi difficiles à convaincre pour la réalisation effective de la réforme, je suis d'ailleurs observé qu'un certain nombre de ces femmes. 2 heures de prolongation sont liés à la réunion d'organismes consultatifs qui ont la vertu de représenter les corps intermédiaires, donc la critique a parfois été fait à l'exécutif de négliger les corps intermédiaires, quand on passe du temps à les écouter, ça justifie d'autres critiques, ça fait partie de la biodiversité politique sur les ordonnances je voudrais terminer en rappelant que c'est une concrétisation importante de la Constitution de 1958 et dans ma mémoire, personne au code et majorité qui se sont succédés depuis 61 ans n'a proposé d'abroger cet article de la Constitution, c'est parce qu'il est bien utile. Il est vrai que ce qu'on renvoie en ordonnance et souvent soit de la législation très complexe, avec d'ailleurs des points de contact dans l'arrêt de législation européenne, ce qui est pas un facteur d'accélération. Et que on renvoie aussi au nord de 11 des choses qui ne sont pas encore prêtes, d'où d'ailleurs, enfin, pour les gens qui ont un peu l'expérience de ça une négociation complexe sur la durée de l'habitation, donc moi j'ai vu plus d'une fois des projets d'ordonnance échoué parce qu'on avait dépassé le délai de d'habilitation, lequel avait été imprudemment fixé trop court, il me semble donc qu'il y a une accoutumance à se donner pour le travail coopératif entre le le le l'exécutif et le législatif sur ce point, je souligne que Luc, les gouvernements successifs et le présent n'y fait pas exception, Monsieur le Ministre, nous jamais proposé de méthode organisé de concertation avec le Parlement pendant l'élaboration des ordonnances.

qui est très observé désormais qui peut susciter autant d'inquiétudes que la phase législative elle-même et parfois plus que des inquiétudes et donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de le faire. Même si ça n'est pas la phase législative elle-même avec un important c'est qu'il faut le faire le le prendre le soin, vous l'avez rappelé d'ailleurs aussi le pouvoir consulter un certain nombre d'organismes qui peut être consultée dans cette phase réglementaire, ça nécessite aussi de veiller, quand même, et tout le monde l'a rappelé à respecter les délais et puis respectez aussi, certains l'ont rappelé ici ce matin, l'esprit de la loi et c'est à ce à quoi nous essayons de nous conformer.

de la constitution, dès 1958 ce gouvernement procède aux ordonnances comme les précédents gouvernements et je crois que celui-là comme les précédents d'ailleurs ont respecté l'esprit de ces ordonnances, c'est ce à quoi il faut veiller, me semble-t-il, ces dispositions qui reste utile qui ont été prévues, je le répète, dès 1958 ce qu'il faut s'éveiller à qui s'essayer de faire en sorte que les équilibres soient tenus et que l'esprit de l'eau, du recours à l'ordonnance soit préservée, maintenue. Merci, la parole est à notre collègue Josiane Costes pour le Rassemblement démocratique et social européen. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues de depuis 1972 le Sénat a inscrit dans son règlement, un dispositif au terme duquel chaque président de commission Grèce annuellement, bilan de l'application des lois leur relevant de la compétence de sa commission en outre sous l'égide du bureau du Sénat un bilan est publié chaque semestre, cela témoigne de l'importance qu'accorde notre assemblée à cette question qu'elle considère comme un impératif démocratique depuis plusieurs années le taux d'application des lois étant mettent hausse conséquence il est vrai, de l'effort du gouvernement en la matière, l'année passée, ce taux était de 73 pourcent, passer à 85 pourcent et le délai moyen de prise des décrets pour les lois votées était d'environ 5 mois cependant, plus de 30 pourcent des décrets étaient pris plus de 6 mois après la boue promulgation de la loi, ces chiffres, bien qu'il soit meilleur que les années précédentes ne peuvent nous satisfaire, dans une période marquée par une défiance des Français envers le pouvoir politique, il est nécessaire de tout mettre en place pour accélérer les effets des textes législatifs afin que nos concitoyens ressentent concrètement les effets des mesures que nous prenons cela passe évidemment par la prise des décrets d'applications, mais également par une coopération de tous les acteurs publics, gouvernements, élus et préfets en 2010, le groupe RDSE avait déposé une proposition de loi tendant à reconnaître une présomption d'intérêt à agir, des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, en matière de recours pour excès de pouvoir, notamment dans le cas où l'exécutif ne prend pas les mesures réglementaires nécessaires dans un délai raisonnable rampante de fait la loi inapplicable, il est souhaitable de remède ce sujet sur la table dans le cadre des débats sur la réforme constitutionnelle S. envisagée, monsieur le Ministre, la crise de la représentativité que traverse notre République n'est pas une fatalité, un des moyens d'y remédier passe par une meilleure application de nos lois sur le territoire, je vous remercie. monsieur le Ministre, les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, il reconnaît bien volontiers que les destinataires de la loi puisse contester le refus d'édicter des mesures d'application et accepte également d'ordonner sous astreinte l'édiction des décrets dans un délai de 6 mois, je crois qu'il avait d'ailleurs été évoquée l'an dernier au sujet de la loi Grenelle 2 en revanche et de jurisprudence constante, le Conseil d'État a fermé cette voie de droit aux parlementaires, ainsi a-t-il rejeté le 23 novembre 2011 le recours formé par le sénateur Masson estimant qu'un parlementaire qui forme un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicite de prendre un décret d'application de la loi ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, le rapport du groupe du Sénat sur la révision de la Constitution, puisque du de ce fait, du coup c'est d'ordre constitutionnel propose de reconnaître au président des assemblées et à 60 députés ou sénateurs, un intérêt à agir pour contester le refus de prendre un décret ça participe du débat constitutionnel, pas s'absolument convaincu que l'émission de la juridiction administrative dans les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels constitue une évolution positive si tant d'ailleurs qu'elle soit nécessaire, le contrôle politique exercé par les assemblées sur l'pourra exécutif a démontré son efficacité nous en donnons un exemple ce matin dans le domaine de l'application des là puisque plus de 90 plus pourcent des mesures d'application des lois sont prises dans les délais, c'est ce contrôle politique que vous exercez en continu et au travers de ce débat annuel qui me paraît devoir être privilégiée à une régulation juridictionnel les désaccords persistants trouveront-ils leur solution dans les mécanismes de contrôle et de responsabilité prévue par la Constit. Communiste républicain et écologiste. Merci monsieur le président me bonjour monsieur le ministre, j'aimerais vous consulter sur la loi 1200 de relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dont l'ambition revendiquée par votre gouvernement, je vous cite était d'agir sur l'écosystème numérique lors d'une campagne électorale nationale comme celle que nous venons de vivre avant les élections européennes, nos 2 commissions avait douté douté de la nécessité la praticité bénéfice de ce dispositif et avait posé par 2 fois la question préalable que le Sénat avait voté dans une très large majorité aussi, je me permets de revenir vers vous pour vous demander comment cette loi été abdiquer lors de cette élection nationale, la prochaine étant l'élection présidentielle, il est vrai, monsieur le ministre, que la loi a été promulguée le 22 décembre 2018 et je comprendrais parfaitement que vous n'ayez pas les informations pour ma réponse mais je, je vous reposerai la question l'année prochaine, donc ça les fera au moins un an avant, service à vos services pour vous renseigner sur le fond, merci. Bien, monsieur le ministre, de toute façon vous dire passerait l'année prochaine. Mais j'espère, avez-vous des éléments, j'espère, monsieur le président, mais dans le cas de la continuité. Le toute façon quelqu'un viendra la continuité sera assurée, c'est pas pour échapper à votre question, monsieur le sénateur, pour tout vous dire, on est dans le domaine de l'application des lois et est-ce le chant qui couvert n'est pas le Champ temporel que celui qu'on vient de puisque le la loi a été promulguée le 22 décembre et dont on est dans le délai de moins de 6 mois, en revanche, ce que je peux vous répondre, c'est vrai qu'on est un peu court en délai mais je peux essayer de regarder quels sont les éléments d'application, là on est sur le, on n'est pas tant sur l'application de la loi sur son utilité, son efficacité, on n'a pas d'éléments, reconnaissons que les élections européennes sont assez récente et qu'on n'a pas d'éléments de recul sur la manière dont les choses ont pu être mises en haut, mais je m'engage devant vous essayer d'obtenir des éléments pour pouvoir voulait transmettre à cette date, c'est difficile de le faire. Merci, Monsieur le Ministre, donner la parole à Franck Menonville le groupe, les indépendants, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le temps de l'application des lois est un temps particulièrement nécessaire au bon fonctionnement de de notre démocratie, il concourt à l'équilibre des pouvoirs, si le Parlement vote les lois, il est crucial qu'ils s'assurent qu'elles sont effectivement appliquées, mais également appliquées conformément au texte qu'il a tout adopter je salue à cet égard le travail remarquable de Valérie Létard et la qualité de son de son rapport qui nous permettent de procéder à cette évaluation suivre l'application des textes votés c'est les qui dit c'est l'exercice du contrôle du pouvoir exécutif, par le Parlement, mais c'est aussi le moyen de s'assurer qu'aucun territoire n'ATT n'a été laissé pour compte, la loi de programmation promulguée le 28 février 2017 et relative à l'égalité réelle outre- mer n'est toujours que partiellement applicable d'ailleurs ce que le président bat également évoqué dans ses propos, le rapport indique ainsi que seuls 16 des 30 mesures d'application prévue par la loi ont été prises en outre trois habilitation à légiférer par ordonnance n'ont pas été suivies d'effet Wallops donc plus de 2 ans que cette loi était promulguée et près de la moitié de ces mesures d'application ne sont toujours pas prises, l'égalité des Outre-mer, avec la peur en métropole est essentiel à l'unité et la cohésion de notre République, monsieur le Ministre, pouvez nous vous nous dire pourquoi, de toutes les mesures d'application de cette loi n'ont pas encore été prise, est ce que vous comptez faire pour y remédier. monsieur le président, monsieur le sénateur Menonville vous avez vous nous interrogez sur l'application de la loi pour l'égalité réelle en outre-mer et vous avez évoqué, c'est vrai, l'utilité de cet échange pour rendre compte de l'application des lois par rapport au chiffre que vous annoncé 4 mesures : l'une à l'article 23 août à l'article 27 sont désormais applicables, ce qui porte à 69 pourcent de taux d'application de ces lois qui est inférieur. à celui du taux d'application pour les autres lois vous avez raison de le signaler. Sur les 9 dernières mesures en attente d'application 3 mesures sont portées par le ministère de la transition écologique et solidaire, article 83 et 138 concernant la mise en place d'un permis chassé en Guyane, le calendrier reste à préciser, sachant que le projet de texte avait fait l'objet d'un avis défavorable du Conseil national de la chasse en octobre 2017 concernant les 2 mesures relatives à l'acquittement d'une redevance pour les centrales géothermiques au profit des communes et des régions sur le territoire desquelles sont implantées, le ministère précise que cette mesure ne pourra être appliqué l'article 138 a omis, en effet, de préciser les modalités de recouvrement qui sont, selon l'article 4 de la Constitution, de nature législative, de plus en métropole, ce dispositif contrevient au mécanisme européen de l'la 6. Sur l'électricité pour y remédier, le ministère envisage d'autres pistes, 3 mesures qui concernent Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont portées par le ministère des solidarités, de la santé qui doit apporter des informations complémentaires sur l'état d'avancement de leur mise en oeuvre et j'y veillerai, le texte consacré à la composition de la commission sur la plus réactivité du comité régional de l'emploi et de la formation et de l'orientation sera publié pour la fin de l'été 2019 la mesure concernant la direction des ressources humaines unique pourrait être prochainement abrogés enfin le projet de loi des chrétiens pro-Latif au fonds de mutualisation et aux modalités d'indemnisation des exploitants agricoles est en cours de préparation cette dernière question, montre bien que l'utilité de cet échange et la nécessité de du travail que vous faites pour. Nous pousser et faire en sorte que nous appliquions mieux les lois qui sont votées, c'est vrai que dans cet exemple là, il y a des Liens encore du chemin à parcourir. Merci monsieur le ministre, 12 acheminons vers la conclusion de notre débat de ce matin, je voudrais d'abord peut-être donner la parole à la présidente Valérie Létard pour qu'on puisse tirer quelques éléments déjà notre échange de ce matin Madame la président. Oui, monsieur le président, et quelques éléments que je souhaitais relevés dans l'ensemble des synthèses qui ont été faits par les présidents de commission et les intervenants peut-être reprendre pour commencer dans l'intervention liminaire de monsieur le ministre, un chiffre qui, quand même, illustre bien les choses entre 2012 et 2018, 346 loi pour 350 ordonnances, ça veut dire qu'un texte sur 2 a fait l'objet d'une ordonnance qui veut dire qu'en clair ça ne permet plus, pour la moitié de ces textes au Parlement de participer de façon satisfaisante à l'élaboration de la loi et on peut considérer que c'est une forme de contournement qui prend de plus en plus d'ampleur et sur lequel nous devons continuer à être attentifs et nous interroger il y a un certain nombre de points récurrent sur ces ordonnances aussi un autre point a été soulevé par les présidents de commission et par exemple celui qui rappelle aussi que les ordonnances, il faut éviter que il s'intéresse à des sujets centraux des textes de loi et que la nature aussi des textes qui font l'objet d'ordonnances doit être regardée avec beaucoup d'attention, il y a eu des points récurrents tels que contrôle des OPEX, le respect aussi de la volonté du législateur dans la prise des textes d'application et vérifier effectivement que de ce point de vue là le législateur soit mieux respectée, un autre point qui rejoint ainsi celui-là le quantitatif ne doit pas cacher le qualitatif et c'est pas parce qu'on a eu beaucoup de décrets d'application beaucoup de textes pris sur Aloise sur une loi sur un texte global qu'il n'y a pas quelques décrets d'application qui sont essentiels au coeur du dispositif d'application de la loi qui n'est pas échapper justement à ces mesures réglementaires en clair c'est pas parce qu'on a un bon taux d'applications qu'on n'a pas pour autant des difficultés à mettre en oeuvre la loi parce que des décrets centraux n'ont pas été pris ou des arrêtés concomitant et j'en conclus en disant que l'utilité de ce travail s'il devait encore, elle devait prouvé, on l'a vu, aujourd'hui elle est avérée, monsieur le ministre nous a rassurés sur des mesures réglementaires qui vont être prises dans les jours qui viennent, d'autres qui viennent d'être prises et on le voit, c'est une saine stimulation de cet échange entre le gouvernement et le Parlement, et nous voulons aussi remercier donc le ministre et le gouvernement de se prêter à cet exercice un petit point si je voudrais rappeler que sur les surtranspositions, il ne faut pas négliger cet aspect et que le travail qui est maintenant par la commission et qui permet de se saisir lorsqu'il y a risque de surtransposition nous apparaît aussi un travail qui peut être très utile en terme de co-élaboration du suivi de l'application de la loi, merci beaucoup. Merci madame la présidente, merci monsieur le ministre, mes chers collègues, l'an prochain. Nous aurons une nouveauté, c'est-à-dire la mise en oeuvre de notre règlement sur le suivi des textes et il faudra bien que nous en fassions aussi une analyse place du rapporteur dans dans le suivi ce des choses j'entendais Alain Richard tout à l'heure et je me suis fait sortir une statistique lors de danse c'est célérité complexité. Si on prend la période 2010 2014, je vais prendre des séquences et la période qui nous sépare 2014, 2017, 2018, 2018 prend pas être pris dans sa totalité parce parce qu'il faudra voir en 2019, il n'empêche que le nombre d'ordonnances en moyenne pondérée sur chacun des séquences quinquennal c'est multiplié par 2. Vous étiez à 27 en 2010, le record c'est 2016 79. Et que cette réalité là il méritera une analyse quand même, je suis trop attaché à la Ve République, je m'exprime Atrides personnel pour dire que l'ordonnance n'aurait pas son utilité, il n'empêche, c'est comme la procédure accélérée, méfions-nous, que ça ne devienne une procédure habituelle et majeur, et je crois que nous serons extrêmement attentifs sur ce point, il y a pas d'hostilité de principe, mais il n'empêche que quand on est multiplié par 2 hommes a une réalité je pense que c'est toute l'utilité aussi que nos débats je voudrais donc vous remercier, remercier particulièrement Valérie Létard parce qu'au-delà de ce rapport annuel et s'est engagé dans ce travail re, vice-président du bureau en charge de ce dossier, je dois vous dire qu'à l'issue de ce débat, nous nous attirons l'attention du 1er ministre généralement lien avec vous, monsieur le ministre, ce que je, je dis : la qualité de nos relations, je le redis publiquement mais je crois que nous avons aussi le devoir d'éclairer le 1er ministre sur l'analyse que nous faisons d'un certain nombre de ces points, on a beaucoup parlé d'ordonnances, il y a aussi des délais, je vois que, parfois, on l'attend les 700 jours on peut se dire qu'on est plus dans l'assiette, mais on est dans le vieillissement pour des cépages qui nécessite un long séjour en feu, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de phénomène d'oxydation, je voulais simplement vous le dire en vous remerciant les uns les autres merci.